La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Dans les régions d'outre-mer, certains produits alimentaires vendus comportent un taux de sucre nettement supérieur à ceux des produits équivalents vendus en métropole. Les industriels justifient cette différence par le fait que le fort taux de sucre permettrait de mieux conserver les aliments. Or, en 2013, la loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer a interdit cette disparité entre les taux de sucre. En effet, la population ultramarine est beaucoup plus touchée par l'obésité que la population hexagonale. pas totalement appliquée par les industriels. Face à l'immobilité des acteurs sur ce problème de santé publique, nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi Lurel et qu'il nous propose des pistes d'amélioration du dispositif.

la fabrication des aliments destinés à nos concitoyens ultramarins. Nous devons avancer sur ces sujets. Le Gouvernement ne

Trop fréquemment, il arrive que les « menus enfants » proposés par les restaurateurs ne soient constitués que d'aliments comportant une forte teneur en graisse : frites, nuggets, steaks hachés.

ou tout autre support, une mention « petit gourmet », laquelle consisterait en un menu contenant au moins un fruit et un légume. Son adoption permettrait, d'une part, d'encourager les parents à veiller sur la qualité nutritionnelle des repas

commission ? C'est une très belle initiative et j'invite les restaurateurs à la mettre en oeuvre. Je ne pense pas pour autant qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi, mais il est certain que cet

38 millions sont en insécurité alimentaire grave, 16 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et, dans notre pays, 4 millions de personnes ont régulièrement recours à l'aide alimentaire.

est à M. le ministre. L'objet de cet amendement est de sécuriser le cadre normatif relatif aux contrôles de l'habilitation des associations au titre de l'aide alimentaire. Un décret concerté devra permettre de clarifier les procédures et les modalités de contrôle qui ne sont pas clairement encadrées par la loi par la loi ou par le règlement. Cet amendement vise à préciser qu'un décret en Conseil d'État détermine non seulement la durée et les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée aux personnes morales pouvant recevoir des contributions publiques destinées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire, mais également les modalités de contrôle de cette habilitation et les sanctions applicables en cas de manquement à ses conditions. Les articles R. 230-10 à R. 230-24 du code rural et de la pêche maritime prévoient déjà les conditions dans lesquelles l'habilitation peut être retirée.

destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire, fondé sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret. Il est préférable de maintenir ces dispositions dans l'article 15, article d'habilitation de ce projet de loi. Le délai de douze mois, prévu pour la publication de l'ordonnance concernée, permettra de mettre en oeuvre les consultations et la concertation nécessaires avec les représentants des collectivités locales, notamment, pour définir précisément les seuils éventuels à partir desquels les opérateurs seraient éligibles et les modalités de mises en oeuvre de ces dispositions visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Quel est l'avis de la commission

cet article prévoit la mise en oeuvre par les gestionnaires de services de restauration collective d'un plan d'action destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire fondé sur un diagnostic préalable avant le 1 septembre 2020. Le Gouvernement a expliqué qu'il convient de mener une concertation, mais rien ne l'empêche de le faire avant de prendre un décret d'application de cet article. En outre, la date de septembre 2020 ne me semble pas très contraignante pour adopter un plan d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire. Avis défavorable. Je mets

Il s'agit en effet de permettre aux élus de prendre en compte ce diagnostic et les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire dans les cahiers des charges qui pourraient être soumis aux gestionnaires de services de restauration publique ou influencer des décisions relatives à l'organisation, aux tarifs, à la composition des repas, aux dépenses de personnel, impactés par ce plan d'action. Par ailleurs, les usagers doivent pouvoir connaître, de la même manière, l'impact de ce diagnostic et du plan de réduction du gaspillage alimentaire sur la qualité des produits, des services, des conditions de prise des repas, ainsi que l'impact budgétaire attendu sur les tarifs.

territoire et du développement durable ? Cet amendement tend à prévoir que le plan d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire mis en place par le gestionnaire de service de restauration collective doit être rendu public auprès des usagers et des assemblées délibérantes. L'article actuel du code de l'environnement qui prévoit une telle démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire par les services de restauration collective gérés par l'État et les collectivités territoriales ne prévoit pas cette publicité. Il ne me semble pas utile d'apporter cette précision dans la loi, qui fixe le principe. Le décret fixera les modalités. Avis défavorable.

mais tous ne se sont pas encore engagés dans la démarche. L'article 15 du projet de loi prévoit déjà de rendre obligatoire pour certains opérateurs de la restauration collective la communication de leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable. Je mets aux voix

sont visés les établissements de restauration commerciale qui proposent une activité de vente à emporter, ainsi que les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter.

Si cette mesure a pu être décriée par certains d'entre vous lors de l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique, nous nous sommes aujourd'hui tous habitués à cette interdiction et nous la saluons. Pendant deux ans, jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure le 1 janvier 2017, les acteurs du secteur ont été accompagnés pour trouver des alternatives au sac plastique à usage unique non compostable ou non biodégradable. Grâce à la recherche et au développement, de nombreuses solutions peu coûteuses existent. Notre amendement est simple, mes chers collègues : il vise à élargir le champ d'application de cette interdiction des sacs plastiques à la restauration de vente à emporter. Pourquoi l'interdire à la distribution, mais l'autoriser au restaurant d'à côté ? Par ailleurs, en cohérence avec l'article 12 A, il serait absurde de pouvoir emporter des aliments non consommés sur place dans un contenant réutilisable, lui-même emballé dans un sac plastique non biodégradable

dans le cadre du programme national nutrition santé. Ces données de santé environnementale en population générale et par publics cibles sont extrêmement importantes et font actuellement défaut. La seule étude consacrée à cet enjeu a été menée par l'Institut national de veille sanitaire en 2006-2007 dans le cadre de l'étude nationale nutrition santé de 2007. Elle avait notamment révélé des concentrations sanguines en polychlorobiphényles chez les Français adultes environ cinq fois plus élevées qu'aux États-Unis et légèrement supérieures à celles observées dans les autres pays européens. noté une moyenne des concentrations urinaires en 2,5-DCP- un chlorophénol - environ dix fois supérieure à celle observée dans la population allemande adulte en 1998, expliquée dans l'étude par une utilisation plus importante de cette substance comme désodorisant ou antimite en France en 2007. Elle avait enfin relevé des concentrations plus élevées en France qu'au Canada et aux États-Unis en pyréthrinoïdes, la famille d'insecticide la plus utilisée en France, tant pour les traitements des cultures que pour les applications domestiques. Le rapport de l'étude cite, par ailleurs, parmi les facteurs influençant les biomarqueurs urinaires le lieu de résidence, notamment la proximité d'une surface agricole dédiée à la culture de la vigne, l'alimentation et l'usage d'insecticides dans le logement. La mise en place d'un système de surveillance de l'imprégnation de la population française par les polluants chimiques, déterminés par les autorités compétentes- l'Institut de veille sanitaire, désormais intégré au sein de l'agence Santé Publique France, l'ANSES, etc. -, englobant les sources de ces polluants, permettrait de collecter les données d'exposition indispensables à la mise en oeuvre d'une réelle politique de santé environnementale.

Cet amendement vise à ajouter au programme national nutrition santé, le PNNS, la mise en place d'un système de surveillance de l'imprégnation de la population par les polluants chimiques. La version actuelle du PNNS, qui couvre la période 2017-2021, comprend des repères nutritionnels à ce sujet, en recommandant une diversification de l'alimentation en faveur de productions moins exposées aux pesticides. Quant à la surveillance de l'exposition de la population aux produits chimiques, elle mérite d'être traitée dans un cadre plus large que les PNNS. En effet, plusieurs points relevés dans l'étude de l'Institut national de veille sanitaire de 2007, citée par les auteurs de cet amendement, ne relèvent pas de l'alimentation, comme la proximité avec une surface agricole traitée avec des produits phytopharmaceutiques ou l'utilisation de produits biocides à l'intérieur du logement. Cette dimension multifactorielle justifie d'avoir une approche globale de l'exposition aux produits chimiques. Sur ce sujet, le troisième Plan national santé environnement prévoit plusieurs actions en complément des mécanismes de surveillance réglementaire existants, notamment sur les résidus de pesticides dans l'alimentation, l'eau potable et l'air.

de l'alimentation, notamment dans l'atelier 8, et d'une thématique qui a fait l'objet de plans d'action de la part de l'État et de ses opérateurs. Le Gouvernement est en train de revoir sa stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Par ailleurs, dans le cadre des études d'alimentation, l'ANSES dresse régulièrement un bilan de l'exposition de la population française, notamment aux substances dites PCB, c'est-à-dire aux polychlorobiphényles. Une nouvelle étude est en cours d'élaboration. Elle fera de nouveau un focus important sur l'ensemble des polluants chimiques. Le souci exprimé à travers cet amendement est parfaitement louable. Il est nécessaire de poursuivre et de renforcer cette surveillance. Nous Nous y travaillons et nous nous y employons. Le PNNS, qui se concentre sur les questions nutritionnelles, n'est pas le bon levier. Il existe, comme je l'ai déjà indiqué par ailleurs, d'autres mesures engagées par l'État et par ses opérateurs. Dans ce contexte, je suis défavorable à l'amendement.

quater La parole est à M. Joël Labbé, sur l'article. Nous arrivons donc au débat sur le bien-être animal. Ce sujet est essentiel, et il faut le traiter sans caricature, mais sans nier non plus les problèmes qui peuvent exister dans ce domaine. Dans les systèmes d'élevages où la logique industrielle est poussée à son comble, l'animal n'est plus considéré comme un être vivant. Il n'est qu'une machine à produire de la viande. J'ai entendu hier, dans cet hémicycle, que, si l'on ne coupait pas les queues des cochons, ils se les mangeaient entre eux.

ce sont bien les conditions d'élevage qui créent ces comportements. On ne peut se cacher ces réalités ! Cela étant, je l'ai déjà dit, je ne remets pas en cause la consommation de viande, je ne prône pas une généralisation du véganisme, même si je respecte le choix de chacun. Je pense que, si un animal d'élevage a eu une vie décente, dans de bonnes conditions, sa mort, son sacrifice pour l'alimentation humaine, car il s'agit bien d'un sacrifice, peut être justifié éthiquement. Pour moi, il s'agit donc de traiter ce sujet en favorisant toutes les mesures qui peuvent permettre d'améliorer le bien-être à la fois des éleveurs et des animaux, et de promouvoir une alimentation durable et de proximité. Les pistes de travail en ce sens sont très nombreuses. Les conditions de vie des animaux sont souvent le reflet des conditions de vie des éleveurs. Je prendrais l'exemple de la qualité de l'air respiré dans les bâtiments d'élevage intensif : cet air où se concentrent des substances nocives est mauvais pour les animaux, qui souffrent d'infections respiratoires. Il est aussi facteur de risque pour la santé des éleveurs. Dans les abattoirs industriels, dénoncés pour les souffrances infligées aux animaux, les travailleurs ne sont pas en reste. Les tâches à effectuer et les cadences sont souvent difficiles ; les maladies professionnelles sont très fréquentes. Si nous favorisons la qualité et la relocalisation de l'élevage, nous favorisons à la fois le bien-être des animaux et celui des éleveurs, qui trouvent une rémunération dans ces systèmes et- ils en témoignent -une fierté retrouvée de leur métier. de leur métier. Les systèmes agricoles qui produisent une alimentation de qualité sont aussi des systèmes où les animaux voient la lumière du jour, ont de l'espace et ont accès à l'extérieur. Sur le volet « mise à mort », si nous favorisons les abattoirs mobiles et les petits abattoirs locaux, nous évitons aux animaux un transport dans des conditions difficiles et une attente dans un lieu inconnu, ainsi que le mélange des troupeaux, qui est source de stress. Je défendrai donc dans ce cadre un certain nombre d'amendements allant dans ce sens. La parole

personne qui a un rapport avec le pays, avec l'environnement sous toutes ses formes, et donc avec le vivant. J'ai connu un temps, pas si lointain, où les éleveurs de la petite région dont je suis originaire donnaient un nom à toutes leurs vaches. Ils amenaient la bête dans la bétaillère avec un sentiment

donc à revenir sur l'extension- à vrai dire assez limitée -du droit des associations de se porter partie civile tel qu'elle est prévue dans cet article. Cela conduirait à abroger tout droit pour ces associations de se porter partie civile dans les cas de maltraitance animale déjà visés par le droit existant.

certaines associations. Je vous invite toutefois à éviter tout excès en la matière. Tout d'abord, l'article 2-13 du code de procédure pénale, dont les grandes lignes datent de 1976, et déjà aux associations de défense et de protection des animaux ainsi qu'aux fondations d'utilité publique de se porter partie civile pour les infractions reconnues dans le code pénal. Le seul apport de l'article 13 du projet de loi consiste à étendre la liste des infractions visées à certaines de celles prévues dans le code rural. Or, s'il pouvait exister une incertitude sur le champ des dispositions visées dans le texte initial, elle a été totalement levée et ce champ a été très très limité par l'Assemblée nationale : seront concernés les seuls délits visés à l'article L. 215-11 dudit code, c'est-à-dire les délits de mauvais traitements qui y figuraient déjà, et qui sont étendus au transport et à l'abattage,

dont le droit de se porter partie civile est reconnu par le code de procédure pénale. Il s'agit en effet d'exiger pour ces associations, et pour elles seules, une reconnaissance d'utilité publique, au lieu d'une simple déclaration régulière depuis au moins cinq ans. Cette dernière condition est exigée pour toutes les associations visées aux articles 2-1 et 2-24 du code de procédure pénale, sur des sujets aussi divers que la lutte contre le racisme, les violences, le harcèlement sexuel, la protection de l'enfance en danger, et bien d'autres.

partie civile sur la base des constats des contrôles officiels. Enfin, nous améliorerons la communication et la formation sur l'expérimentation, par exemple dans le cadre du Conseil national de l'alimentation, de l'étiquetage relatif à l'origine des produits, et sur d'autres marqueurs attendus

de se porter partie civile pour les infractions de maltraitance animale. Je précise d'ailleurs que les associations ne peuvent se porter partie civile que sur la base de contrôles officiels réalisés par des agents formés et assermentés. J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

n'ont jamais été conduits de la même façon selon qu'il s'agissait de bovins lait, de bovins viande, de lapins, de poules, de cochons ... Au Moyen Âge, les porcs vivaient dans des cases, cases, mangeaient beaucoup moins bien qu'aujourd'hui et ne voyaient pas non plus la lumière du jour. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des élevages de porcs en plein air, mais ils ne sont pas très heureux

les quelques excités que vous avez cités n'ont aucune relation avec cette forte baisse de la consommation de viande, qui trouve

de l'alimentation. Est-il logique de transporter pendant plus de douze heures des animaux vivants, alors que nous pouvons relocaliser les productions au bénéfice des consommateurs, de l'environnement, de l'économie locale et des éleveurs ou des paysans ?

européen, lequel ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre, ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre. Par ailleurs, un certain nombre d'États membres demandent à ce que soient renforcées les exigences en matière de limitation de la durée des transports. C'est le cas de l'Allemagne, du Danemark, de la Belgique, des Pays-Bas, qui ont porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016. La France ne sera donc pas isolée si elle adopte une telle position. On parlait précédemment des demandes et des attentes sociétales : cela en fait partie. L'amendement

entre les pays de l'Union européenne et définit les modalités des contrôles opérés à l'entrée ou à la sortie de celle-ci. Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport, mais uniquement des limites de temps de route successifs 29 heures pour les bovins, ovins et caprins, 24 heures pour les chevaux et pour les porcs, 19 heures pour les animaux non sevrés. Au-delà, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos de 24 heures avant de reprendre la route. Chaque État membre de l'Union européenne est soumis à l'application de ce règlement. Cependant, l'article 1 du règlement prévoit que ce dernier « ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre ». Depuis plusieurs années, les ONG de protection des animaux dénoncent régulièrement, en s'appuyant sur des enquêtes détaillées, des conditions de transport non compatibles avec la protection minimale des animaux.

Selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, paru en 2004, après quelques heures le bien-être des animaux se détériore sévèrement. En 2012, le Parlement européen s'était d'ores et déjà prononcé pour une limitation à 8 heures de la durée de transport des animaux destinés à l'abattage, appuyé par une pétition signée par plus d'un million de de citoyens européens. La Fédération des vétérinaires d'Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l'exportation des bovins [ ...] conduisant à la souffrance, l'épuisement et parfois même la mort des animaux appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d'animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant, en conclusion, que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production un certain nombre d'États membres demandent aujourd'hui une révision du règlement n° 1/2005 précité afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C'est ainsi le cas de la Suède, la Suède, appuyée par l'Allemagne, le Danemark, la Belgique, l'Autriche et les Pays-Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016, en affirmant qu'« afin d'améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement n° 1/2005], notamment sur les temps de parcours

pour les transports se déroulant exclusivement sur le territoire français. Or, vous l'avez dit, mes chers collègues, les règles applicables en matière de transport sont harmonisées au niveau européen : elles fixent déjà un certain nombre de prescriptions, qui peuvent toujours paraître insuffisantes aux uns ou aux autres. À titre d'information, les animaux ne peuvent voyager plus de 8 heures, sauf si le moyen de transport remplit toute une série de conditions très très précises. Je rappelle, par ailleurs, que l'article 13 du projet de loi a étendu le délit de maltraitance au transport. Nous avons doublé les sanctions et permis aux associations de se porter partie civile en cas d'infraction

mais je pense aussi au transport d'animaux vivants vers d'autres pays pour lesquels les temps de transport sont un peu plus longs. Il faut bien évidemment prendre toutes les précautions, mais aussi veiller à ne pas tuer des pans entiers de notre économie tournés vers l'exportation ni les grands rassemblements ou rendez-vous comme le Salon de l'agriculture.

traitant de ces questions. Le représentant des transporteurs qui était présent- il était d'ailleurs très intéressant de l'entendre -nous a dit que la réglementation sur le temps de travail des chauffeurs était incompatible avec celle sur le transport des animaux vivants.

tend à introduire un encadrement spécifique des exportations d'animaux vivants vers des pays hors de l'Union européenne, par l'obligation d'introduire dans les accords de partenariat avec les pays de destination des clauses encadrant la protection des animaux dans ces pays, ainsi que la mise en place d'un certificat à l'export sur le modèle australien. En effet, chaque année, environ 3 millions d'animaux sont exportés de l'Union européenne vers des pays tiers, notamment vers l'Afrique et le Moyen-Orient. La France figure parmi les premiers exportateurs, principalement vers les pays d'Afrique du Nord. La réglementation européenne relative à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes s'applique théoriquement aux animaux même lorsqu'ils ont quitté l'Union européenne. Pourtant, une fois franchies les frontières de l'Europe, la réalité est tout autre les voyages peuvent durer jusqu'à 14 jours dans des conditions d'extrême densité de chargement, sous des chaleurs dépassant parfois les 40 degrés, sans temps de repos approprié, ni suffisamment de nourriture ou d'eau ; l'engraissement et l'abattage à l'arrivée se déroulent dans des conditions qui, pour la plupart, sont contraires aux standards internationaux de l'Organisation mondiale de la santé animale, Depuis 2011, à la suite de nombreux scandales relatifs aux conditions de traitement des animaux dans les pays de destination, l'Australie a mis en place un système assurantiel, qui exige des exportateurs de garantir que les animaux seront traités à l'arrivée en conformité avec les recommandations de l'OIE sur le bien-être animal. Le présent amendement s'inspire de l'exemple australien, en prévoyant un encadrement des règles d'exportation des animaux vivants vers des pays hors de l'Union européenne.

hors de l'Union européenne par l'obligation de conclure des accords de partenariat avec les pays de destination et de disposer d'un certificat à l'export, afin de s'assurer de la protection de ces animaux dans ces pays de destination. Là encore, si elle n'est pas négociée dans le cadre d'accords commerciaux multilatéraux, une telle obligation serait particulièrement discriminante pour les seules exportations françaises et, par ailleurs, peu contrôlable. L'avis est donc défavorable.

dans ce domaine, mais elles s'appuient sur plusieurs leviers d'action aux niveaux international et européen. Des dispositifs de communication ont été développés avec des pays tiers, comme Israël, pour échanger sur l'état général des animaux lors du déchargement dans le pays importateur. La France développe de nombreuses coopérations avec les pays tiers pour partager ses expériences dans les domaines de la sécurité sanitaire, de la santé et de la protection animales. Au niveau européen, les autorités françaises veillent à ce que le bien-être animal soit bien couvert dans le cadre des négociations menées par la Commission. S'agissant des accords de libre-échange entre l'Union et les pays tiers, et dans chaque négociation, il s'agit de mettre en place une

Les couvoirs industriels produisent 90 millions de poussins chaque année aux fins de sélectionner des poules de races pondeuses. À l'éclosion, 50 millions d'entre eux s'avèrent être des poussins mâles et sont donc broyés vivants. un arrêté du 12 décembre 1997 autorise l'utilisation de ces dispositifs mécaniques de broyage, il est temps d'affirmer que faire naître des animaux pour les tuer à leur naissance n'est ni éthiquement acceptable ni

rectifié. Nous sommes tous particulièrement mal à l'aise face à ces pratiques, mais il n'existe pas, à ce jour, de méthodes alternatives qui soient parfaitement validées et industrialisables à court terme. Nous sommes néanmoins vigilants

La coupe systématique des queues est déjà interdite par la réglementation communautaire : la section partielle de la queue peut être réalisée, non sur une base de routine, « mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu » et après que d'autres mesures ont été mises en oeuvre. Il est nécessaire de préserver cette possibilité en cas de besoin et de responsabiliser les professionnels sur le cadre strict de la réglementation. J'ai souhaité, dans le droit-fil de la stratégie en faveur du bien-être animal,

? Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes alternatives à la castration à vif des porcelets.

L'utilisation de systèmes d'élevage en cage pour les poules pondeuses est aujourd'hui perçue de façon négative, affaiblissant la confiance des consommateurs dans les filières d'élevage

Un accompagnement financier devra être mis en place, afin de soutenir les producteurs dans cette évolution de leurs systèmes d'élevage. Quel est l'avis de la commission ?

Cela permettra notamment que la totalité des oeufs coquilles vendus aux consommateurs soient issus de volailles élevées dans le cadre desdits systèmes de production alternatifs à la cage. À cet effet, l'article 13 A prévoit que tout nouveau bâtiment

la réglementation européenne avait évolué, à la suite d'une demande très forte de faire agrandir les cages, justement au regard de cette question du bien-être animal. L'ensemble des exploitants ayant ainsi

Les consommateurs n'achètent plus les autres parce que, quand ils consomment un oeuf, ils ont en tête la malheureuse poule dans sa cage, ce qui les bloque.

De temps en temps, il y a donc des combats d'arrière-garde qui ne méritent pas d'être menés ; il faut adapter les méthodes et écouter un peu les consommateurs parce que de toute façon,, ce sont eux qui décideront.

? Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui a réintroduit dans le texte la possibilité de réaménagements ; il n'y a pas lieu d'interdire tout réaménagement d'un bâtiment existant.

qu'un producteur soit amené à faire des aménagements accessoires, mais bénéfiques aux animaux. En pratique, le recentrage de l'interdiction sur les bâtiments nouveaux n'affaiblit nullement la portée dès lors que, au vu des perspectives de marché, aucun producteur ne trouverait aujourd'hui un intérêt économique à réaménager son bâtiment dans l'objectif, non pas de répondre à une difficulté ponctuelle ou d'améliorer le bien-être des animaux, mais d'augmenter sa production d'oeufs en cage ou de démarrer une nouvelle production. Il s'agit donc

donc un avis défavorable sur ces amendements

dites, monsieur le ministre, que la chose est réglée avec la filière et que l'objectif est de faire disparaître ce mode d'élevage, j'entends cet engagement.

très consensuels dans ce débat sur le bien-être animal. Je n'ai pas souhaité m'exprimer plus tôt sur les autres sujets, j'ai voté comme la commission et comme le ministre sur tous les amendements, mais il me semble que, sur ceux-ci, il faut y réfléchir un peu, car cela vaut la peine d'envoyer ce signal.

Cet amendement tend à interdire progressivement l'élevage des lapins en cage. En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées, où l'espace de vie est très restreint- l'équivalent d'une feuille de format A4 par lapin source de stress, d'inconfort permanent et de blessures, empêchant l'expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux. La hauteur des cages utilisées est ainsi insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière. Un avis scientifique portant sur l'influence des systèmes actuels de logement et d'élevage sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d'élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a mis en lumière les nombreux problèmes de bien-être animal et de santé qui y sont observés. L'EFSA souligne en effet que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement hauts, en raison d'une forte exposition aux maladies parasitaires. Plus de dix ans plus tard, les mêmes problèmes perdurent et aucune mesure n'a été prise pour y remédier. La France, qui est le deuxième pays européen producteur de lapins élevés pour leur viande, ne dispose d'aucune législation sur le bien-être des lapins, contrairement à d'autres pays européens, comme la Belgique, qui interdit l'utilisation de cages, ou l'Allemagne et l'Autriche, qui définissent des standards minimaux. En mars 2017, le Parlement européen a d'ailleurs adopté une résolution sur l'adoption de normes minimales relatives à la protection des lapins d'élevage, encourageant les éleveurs de lapins à éliminer les cages. Cet amendement vise donc à mettre en place des standards minimaux de bien-être des animaux en élevage cunicole, en incluant l'interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parcs collectifs enrichis à compter du 1 janvier 2025 pour les lapins d'engraissement, et du 1 janvier 2030 pour les reproducteurs et le précheptel.

Alors que la consommation de viande de lapin ne cesse de baisser, un mode d'élevage plus conforme au bien-être animal serait de nature à rassurer le consommateur et à favoriser la filière cunicole.

La commission propose, plutôt que de procéder par interdiction, de faire confiance aux filières, qui ont pris des engagements forts en la matière. Je le rappelle, le plan de la filière cunicole pour la période 2018-2022 s'engage à faire passer de 1 % à une

à trouver, à travailler. Nous suivons cela de près. Un travail est mené par convention avec un institut technique pour déterminer ce qui serait le bâtiment du futur pour les lapins.

où se mouvoir. Ce travail est en cours. Le Gouvernement est soucieux de cette évolution et espère que l'on pourra déterminer le meilleur système

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le respect du bien-être animal est un sujet important de préoccupation, notamment pour nos concitoyens. Bien qu'elle soit très clivante, je pense que nous devons aborder cette question avec pragmatisme et sans aucun dogmatisme. C'est pourquoi je regrette que le bien-être animal ne soit pas considéré dans toutes les filières, En effet, l'article 13 prévoit de faire évaluer les réalisations concrètes en matière d'amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés par les plans de filière des organisations interprofessionnelles. Pourtant, le pastoralisme est exclu de ce dispositif, puisque la souffrance occasionnée par les attaques de loups sur les animaux d'élevage n'est pas prise en compte par le projet de loi. En application de l'article L. 214-5 du code rural et de la pêche maritime, un centre national de référence sur le bien-être animal a été créé le 28 février 2017. J'ai déposé récemment un amendement, qui a été déclaré irrecevable, tendant à demander une expertise technique sur l'impact de la prédation et des mesures de protection sur le bien-être des animaux d'élevage. En effet, à titre d'exemple, le nombre d'avortements enregistrés par les éleveurs sur les brebis prédatées est très significatif. Les animaux qui survivent sont en réelle souffrance, et je regrette que cette souffrance animale ne suscite pas le même intérêt que d'autres.

Le présent amendement est important ; il vise à préciser que le rapport attendu du Gouvernement porte sur l'adéquation entre les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes en matière de bien-être animal prévues dans les plans de filière élaborés par les organisations interprofessionnelles à l'issue des Il nous faut évidemment évaluer les actions conduites par les filières en matière de bien-être animal, au regard des attentes sociétales telles qu'elles se sont exprimées au cours des États généraux de l'alimentation. Quel est l'avis de la commission ?

Le règlement n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l'Union européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l'entrée ou à la sortie de l'Union européenne. Chaque État membre de l'UE est soumis à l'application de ce règlement ; cependant, l'article 1 du règlement prévoit qu'il « ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre Les conditions de transport maritime sont aujourd'hui insuffisamment encadrées par la réglementation européenne, qui ne comporte que peu de dispositions spécifiques au transport maritime. Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2017 par l'ONG faisait état d'infractions importantes et régulières à la réglementation, en particulier en raison de l'absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection. Afin d'y remédier, et à l'instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du règlement n° 1099/2009, cet amendement vise à mettre en place un responsable de la protection des animaux sur les navires bétaillers.

navires bétaillers. Le règlement européen du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l'Union et définit les modalités de contrôles opérés à l'entrée ou à la sortie de l'Union européenne. Chaque État membre de l'Union européenne est soumis à l'application de ce règlement. Cependant, l'article 1 du règlement prévoit qu'il « ne fait pas obstacle à d'éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d'un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d'un État membre ». Les conditions de transport maritime sont aujourd'hui insuffisamment encadrées par le règlement européen, qui ne comporte que peu de dispositions spécifiques au transport maritime. Or de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Afin d'y remédier, et à l'instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du règlement n° 1099/2009,

En visant les navires au départ du territoire français, la contrainte pénaliserait prioritairement les navires français et l'exportation d'animaux issus d'élevages français. Et qu'adviendrait-il, mes chers collègues, de l'autorité du responsable de la protection des animaux, dont on nous dit qu'il serait indépendant,

Quel est l'avis du Gouvernement ? des animaux durant le transport. Les autorités françaises s'emploient à rechercher des modalités pratiques de mise en oeuvre des formations prévues pour les équipages des navires et les dockers dans les ports de chargement. Légiférer au sujet de la désignation d'un RPA

Il semble pour le moins préjudiciable et aberrant que, pour des opérateurs exerçant aux postes d'abattage, l'obtention d'un certificat d'aptitude, pourtant prévue par la réglementation, ne soit pas, encore aujourd'hui, effectivement exigée. À ce défaut courant de formation initiale s'ajoute l'absence de formation continue. Pourtant, le règlement européen n° 1099/2009 du 24 septembre 2009, entré en vigueur en France le 1janvier 2013, recommandait la délivrance d'un certificat de compétence en matière de protection animale pour les opérateurs chargés de la mise à mort en abattoir. Or, cinq ans après, il est toujours très mal appliqué, à la faveur d'un régime transitoire d'application instauré pour permettre l'adaptation des exploitants des établissements. En effet, de nombreux opérateurs sur la chaîne de mise à mort exercent cette mission délicate sans être titulaires

À l'opposé des sacrificateurs procédant à l'abattage rituel, qui, eux, se voient imposer une certification obligatoire, il est urgent, au vu des scandales qui ont éclaté récemment, que l'on impose un délai de régularisation pour satisfaire à cette obligation de bon sens. La vérification de la validation de la formation requise, puis la charge d'une formation continue

La commission entend vos arguments avec une certaine surprise puisque, officiellement, ces personnels doivent disposer d'un certificat attestant de leur compétence, de leurs connaissances au regard du respect de la réglementation en matière de protection des animaux. Ce certificat, intitulé « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort », est délivré par le préfet, sous réserve du respect d'exigences en matière de formation et de réussite à une évaluation.

Toutes les investigations montrent les conditions de travail extrêmement difficiles dans les abattoirs, en particulier aux postes de saignée. Il faut l'admettre, peu de personnes accepteraient de travailler dans de telles conditions, pour une telle activité. Comment le nier ? Nous mangeons de la viande, pour ceux qui en mangent encore, mais peu d'entre nous supporteraient d'abattre des animaux huit heures par jour. Ce sont là des conditions extrêmes. Accuser les individus qui dérapent sans remettre en cause le système ne changera pas les choses pour les animaux. Dans les abattoirs, les deux souffrances, animale et humaine, sont liées. Il faut évidemment travailler sur les conditions de travail, la formation, la réduction des cadences. des cadences. Un journaliste d'investigation ayant passé six mois dans un abattoir a souligné que 30 % à 40 % des effectifs pour les saignées sont composés d'intérimaires et que la formation est absolument inexistante.

devons y réfléchir. Quel est l'avis de la commission ? La commission est favorable à une expérimentation de la vidéosurveillance, mais sur la base du volontariat, avec l'accord des salariés et de l'exploitant. Cette expérimentation nous semble plus équilibrée et respectueuse de l'ensemble des droits

Donc, accompagner, c'est former les gens qui travaillent dans les abattoirs à ces postes difficiles à faire le meilleur geste possible, celui qui occasionnera le moins de souffrance à l'animal.

: La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue. Cet amendement tend à mettre en oeuvre un engagement présidentiel. La révélation de cas de maltraitance animale a jeté le discrédit sur les 263 abattoirs que compte la France. Il s'agit aujourd'hui de redonner confiance aux éleveurs et aux consommateurs dans la filière d'abattage. Il s'agit également de permettre aux salariés des établissements d'abattage de travailler dans de bonnes conditions et d'être fiers du travail qu'ils accomplissent. Cela fait plusieurs années que le Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire préconise le renforcement des contrôles et la mise en place de caméras au niveau des postes de saignée. La mise en place de la vidéosurveillance poursuit un triple objectif : la prévention, la formation et la répression. S'il est difficile de qualifier la souffrance animale sur la base de vidéos, il est en revanche aisé de mettre en lumière une mauvaise pratique d'abattage ou un comportement maltraitant. Il s'agit d'évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal. Aussi, en proposant une expérimentation, l'article 13 A va indubitablement dans le bon sens. L'argument du Big Brother n'est pas sérieux. Cette expérimentation sera en effet réalisée sous le contrôle de la CNIL, qui n'autorise pas que les salariés soient sous surveillance permanente ou constante. En revanche, on ne peut se satisfaire d'une expérimentation sur la base du volontariat sans aucune solution de repli. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que cette expérimentation sera réalisée dans un établissement d'abattage par département, sur la base du volontariat ou, à défaut, par tirage au sort.

pervers serait que les dirigeants de l'abattoir puissent ainsi surveiller leurs salariés en permanence.

? Le recours au tirage au sort est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé de porter à la connaissance des consommateurs les dispositifs de contrôle interne

n° 549 rectifié, les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation seront définies par décret, après un avis de la CNIL. Elles préciseront les modalités de recueil de l'avis des institutions représentatives du personnel. L'ajout proposé n'est pas du domaine de la loi.

? Ces amendements visent à étendre l'expérimentation prévue pour les abattoirs mobiles aux petits abattoirs non mobiles dans les zones non pourvues d'un abattoir de proximité ou qui sont mal desservies. La commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une telle extension, qui pourrait être intéressante,

toute la nomenclature et les mesures environnementales et sanitaires nécessaires pour un abattoir. En effet, nous devons bien évidemment rester très attentifs à la sécurité sanitaire des aliments que consomment nos concitoyens.

la collectivité a fait le choix de racheter le foncier et l'immobilier et d'engager sa modernisation et sa mise aux normes,

Toutefois, nous estimons aussi que la création de structures mobiles pourrait fragiliser les abattoirs de proximité existants. La rédaction actuelle de cet article 13 prévoit que cette expérimentation se traduira par une évaluation de la viabilité économique et de l'impact sur le bien-être animal de ces unités mobiles.

jours ouvrés, plutôt que 365 jours par an. Les accidents touchent chaque année de nombreux animaux d'élevage, sans aucun lien avec la maltraitance animale. Selon Interbev, 50 000 bovins sont accidentés chaque année dans les élevages français. La prise en charge rapide des animaux accidentés est nécessaire pour plusieurs raisons : ne pas causer de souffrance inutile aux animaux ; limiter les risques sanitaires, l'allongement des délais d'attente pouvant se matérialiser par de la fièvre ou une propagation des lésions ; se placer dans un souci de réduction du gaspillage alimentaire, les animaux non pris en charge quarante-huit heures après l'accident ne pouvant réglementairement plus être abattus en vue d'une commercialisation de leur viande. Or les abattoirs reçoivent les animaux accidentés transportables et les carcasses d'animaux accidentés non transportables sur une base volontaire. Cette activité étant peu rentable pour eux, elle est de moins en moins proposée aux éleveurs. Les délais d'attente des animaux en ferme et le risque de non-prise en charge des animaux accidentés s'accroissent donc au fur et à mesure que ces services disparaissent. Il convient donc de les remettre en place.

animaux accidentés transportables. Il vient répondre à une attente forte du monde agricole, car le nombre de bêtes perdues chaque année du fait de l'absence de ce type de service est de plus en plus important. Selon l'interprofession, 50 000 bovins sont accidentés annuellement.

pourra fixer la liste des destinataires de ces informations et la fréquence de leur envoi. Ces informations pourront servir de base aux discussions entre abattoirs, éleveurs, clients, État et collectivités, par exemple lors des groupes locaux de concertation et de dialogue sur les abattoirs-

Madame la ministre, mes chers collègues, aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la Constitution, « le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin Je vais lever la dernière séance de la session ordinaire, qui sera close samedi 30 juin à minuit. À partir du lundi 2 juillet, le Parlement sera réuni en session extraordinaire.

la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous